J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque le texte adopté par l'Assemblée nationale nous a été transmis en février dernier, un accord en commission mixte paritaire était loin d'être une évidence, tant les sujets de désaccord entre nos deux assemblées étaient nombreux.

néanmoins que cet accord est un bon accord, en premier lieu parce qu'il est favorable à l'école de la République, à ceux qu'elle sert et à ceux qui la servent. Sans esprit de parti, ou- devrais-je dire -d'assemblée, l'aspect positif de ce compromis tient en ce qu'il reprend une grande partie des apports du Sénat. La Haute Assemblée a ainsi apposé son empreinte sur ce projet de loi, autour de trois axes : le retour aux fondamentaux de l'école, la prise en compte des réalités locales et des collectivités territoriales et, enfin, l'ambition d'une transformation profonde de notre système éducatif.

qui, tout en rappelant l'exigence d'exemplarité des professeurs, met celle-ci au service de leur autorité et inscrit clairement le respect dû par les élèves et leur famille aux professeurs dans les fondements du code de l'éducation.

de l'école. Les comportements portant atteinte à la liberté de conscience des élèves ont été interdits dans l'enceinte des établissements scolaires, mais également aux abords immédiats de ces réaffirmées, avec le renforcement du contrôle de l'instruction en famille et de l'enseignement privé hors contrat, tout en donnant les garanties nécessaires à l'exercice de la liberté de l'enseignement. Cette ambition s'est également traduite par le renforcement du volet consacré à l'école inclusive, qui désormais est aussi un principe fondamental de l'école, un principe à l'élaboration duquel le Sénat a pris toute sa part. nous avons retenue, rôle constitutionnel du Sénat oblige, fut de prendre en compte les réalités locales. Nous avons donc consulté et entendu les élus locaux. Aussi, nous avons supprimé définitivement l'article 6 et avons inscrit les clarifications nécessaires pour garantir l'accueil des enfants de 3 à 6 ans dans les écoles à classe unique. De même, nous avons enregistré la possibilité de déroger, dans un cadre contractuel, à l'obligation d'assiduité en petite section. Introduite par le Sénat, cette disposition a été maintenue dans le texte de la commission mixte paritaire, et je m'en réjouis.

Tout simplement parce que depuis soixante-dix ans, les maires ont porté l'ambition d'une école maternelle ouverte à tous et qu'ils ont ainsi couvert la France d'un blanc manteau d'écoles maternelles Il fallait saluer cette volonté qu'aucune loi n'obligeait et qui inscrit notre pays parmi ceux où l'obligation d'instruction est la plus précoce. Mes chers collègues, soyons fiers du travail des maires ! Soyons également fiers d'avoir oeuvré collectivement pour abaisser à 3 ans l'âge de la scolarisation obligatoire et d'avoir adopté cette disposition à l'unanimité Le Sénat a porté l'ambition d'une évolution profonde du système éducatif, dont les principaux leviers sont l'expérimentation, l'évaluation et la formation des enseignants.

et la possibilité de déroger, dans le cadre de ces expérimentations, aux obligations réglementaires de service des enseignants. Deuxièmement, a été fixée une nouvelle composition du Conseil d'évaluation de l'école, garante d'une indépendance accrue. entériné l'enrichissement du contenu de la formation initiale des enseignants, notamment au regard des enjeux du développement durable, du numérique, chère présidente Catherine Morin-Desailly, et des spécificités ultramarines. été retenues l'introduction d'une formation complémentaire des enseignants pendant les trois ans suivant leur formation initiale et l'inscription du caractère obligatoire de la formation continue pour tous les enseignants. Ce sont là des apports majeurs du Sénat. tous ces apports, que j'estime, je le répète, importants, ont été sauvegardés au prix de concessions sur des points du texte qui nous tenaient pourtant à coeur. Je citerai : la possibilité de sanctionner les manquements à l'obligation d'assiduité par la suppression des allocations familiales l'application du principe de neutralité aux accompagnants de sorties scolaires ; l'autorité hiérarchique du directeur d'école ; l'affectation sur contrat de mission ; l'avis du chef d'établissement pour les affectations. Autant de sujets dont nous aurons à reparler. Deux points, surtout, constituent à mes yeux des concessions majeures. D'une part, les jardins d'enfants devaient disparaître, mais nous avons obtenu l'allongement de deux à cinq ans de la dérogation accordée à ces structures, afin qu'elles accueillent des enfants de 3 à 6 ans. Ce délai devrait faciliter leur reconversion en école hors contrat,

surtout, nous avons dû céder sur la compensation des communes qui jusqu'alors participaient au financement des classes maternelles privées sous contrat, sans toutefois verser la totalité de la somme correspondant au coût d'un élève dans le public. Le Sénat avait clairement pris position sur le sujet, en l'inscrivant à l'article 4, considérant que l'absence d'une telle compensation, si elle pouvait se justifier sur le plan juridique, n'en constituait pas moins une injustice. Le Gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale sont restés sourds à nos arguments, je le regrette. Il leur reviendra de prendre leurs responsabilités. Pour notre part, nous demeurerons vigilants quant aux modalités de compensation et aux conséquences de l'instruction obligatoire dès 3 ans sur les finances des collectivités territoriales. Ces concessions, pour lourdes soient-elles, ne doivent pas nous faire oublier tout ce que le Sénat a obtenu et que j'ai rappelé au début de mon propos. C'est pourquoi en conscience, mes chers collègues, je vous invite à adopter le texte qui nous est soumis aujourd'hui.

Ce consensus fondateur donne un rôle majeur à l'école, celui de compenser les inégalités. Espérons que l'effort porté sur l'école maternelle comme lieu des premiers apprentissages- effort qui sous-tend ce texte -confortera cette mission première de notre école. Ce consensus fondateur fait aussi de l'école le creuset de l'équité territoriale. Nos débats ont montré l'attachement des élus et des familles à cette « école de la proximité », qui, partout dans le pays, donne une chance à tous.

confiance dans la société qui les missionne. Certes du chemin reste encore à parcourir sur le sujet, mais la volonté est partagée. Oui, mes chers collègues, l'école peut nous rassembler, pour que nous fassions autour d'elle République

d'une confiance renouvelée en la promesse scolaire, en la promesse républicaine de progrès et de justice sociale. Le projet de loi soumis par le Gouvernement s'articulait autour de deux axes.

d'amendements adoptés, le travail parlementaire a permis à la fois d'améliorer le projet de loi initial soumis par le Gouvernement et de l'étoffer avec des dispositions essentielles. Je pense tout d'abord à l'école inclusive- j'y ai déjà fait référence -qui fait l'objet d'un nouveau chapitre entier de ce texte. Ces dispositions entreront en vigueur dès la rentrée de 2019 et permettront une transformation copernicienne de nos organisations, pour faire émerger un grand service public du handicap inédit à l'école.

du texte : la formation continuée, le renforcement de la formation continue, ou encore l'enrichissement du contenu de la formation initiale des professeurs. Ces nouvelles dispositions complètent les dispositions initiales de ce projet de loi relatives à la création de ce que nous appelons désormais les Le rapport de la présidente de la commission de la culture, Mme Catherine Morin-Desailly, a permis d'enrichir la formation initiale des professeurs dans le domaine du numérique, et je l'en remercie. Je souhaite aussi rendre hommage aux propositions de loi, déposées notamment par les groupes communistes et socialistes, qui visaient à abaisser l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. J'ai plusieurs fois indiqué que cet enjeu, que ces groupes

Je pense enfin à tous les sujets ayant émergé grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, au cours du débat parlementaire. Ils se nourrissent de vos sensibilités politiques et de vos expériences d'élus de terrain. Je citerai l'assouplissement des conditions d'assiduité en petite section de maternelle ; le renforcement de l'indépendance du futur conseil d'évaluation de l'école l'amélioration des garanties de mixité sociale au sein des EPLEI ; la création de dispositions législatives spécifiques pour lutter contre le harcèlement à l'école ; les jardins d'enfants qui bénéficieront d'une période dérogatoire et dont nous devons garder toutes les caractéristiques

Je pense également au travail partenarial qui sera engagé avec les collectivités territoriales, notamment sur les décrets d'application et le projet d'ordonnance. Je pense aussi à tous les chantiers que nos discussions

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme d'un insoutenable suspens, la droite ... et la droite se sont donc mises d'accord sur un projet commun pour notre école

362 écoles qui vont être fermées. Aucune sans l'accord du maire, a indiqué le Président de la République à l'issue du grand débat ... Mais à force de diminutions de dotations, de pressions, pas toujours amicales, en faveur de regroupements d'écoles, de nombreux maires se résignent à la fermeture. D'autres doivent recourir à la justice pour se faire entendre. Vous sembliez pourtant convenir lorsque nous avions abordé le sujet, monsieur le ministre, de la nécessité de renforcer le dialogue, afin de ne pas en arriver à cette judiciarisation, qui n'est bonne pour personne. Sous cet angle, il reste des marges de progrès. Certes, ce mouvement n'est malheureusement pas nouveau- l'Association des maires ruraux de France montre que, depuis le début des années 1980, le nombre d'écoles a diminué quatre fois plus vite que le nombre d'enfants. fait devient de plus en plus insupportable à mesure que nos concitoyens voient leur territoire abandonné par la plupart des services publics et des institutions républicaines. Dans ce contexte, nous nous réjouissons, et c'est bien là la seule vraie victoire pour nos territoires et nos enfants, que la forte mobilisation ait eu raison des établissements publics des savoirs fondamentaux, comme notre assemblée l'a souhaité. Ces derniers auraient effectivement accéléré cet affaiblissement du service public de l'éducation dans nos territoires. Aux côtés de toute la communauté éducative, des élus et des parents d'élèves, nous resterons extrêmement vigilants sur ce point. Contrairement aux annonces du Président de la République, là encore à l'issue du grand débat, la généralisation de classes à moins de 24 élèves en grande section de maternelle, cours préparatoire- pour cette rentrée. Dans l'académie de Rouen, par exemple, vos services sont en train de réexaminer- je souhaite vivement que des postes soient attribués - la situation de classes de maternelle à plus de 30 élèves De tels effectifs en maternelle affaiblissent la mesure que vous vouliez « phare » de ce projet de loi. Pour que l'instruction obligatoire à partir de 3 ans soit le progrès social que vous revendiquez, et que nous défendons pour notre part depuis toujours, alors il faut garantir un bon accueil des plus jeunes enfants

le nombre de postes ouverts au dernier concours de professeurs des écoles a diminué de 45 unités par rapport à l'an passé. Ce n'est évidemment pas un cas isolé ! Cette réduction du nombre de postes ouverts au concours se conjugue à une nette dégradation de l'attractivité du métier d'enseignant. Au plan national, ce sont plus de 800 postes qui risquent de ne pas être pourvus à la rentrée. C'est davantage qu'en 2018, où leur nombre était déjà supérieur à celui de 2017. Voilà pourquoi aucune de nos craintes n'est véritablement levée sur le sort des assistants d'éducation, qui ne sont plus garantis, à l'issue de la commission mixte paritaire, de disposer d'un enseignant-tuteur. Dans un contexte de pénurie organisée, le risque est grand qu'ils ne se retrouvent devant des classes. Si la formation continue des enseignants hors temps de travail a été supprimée du texte issu des travaux du Sénat, vous avez publié un décret, monsieur le ministre, permettant de réquisitionner les enseignants sur leur temps de vacances. S'agissant de l'école inclusive, j'ai déjà eu l'occasion de dire nos craintes que ne se substituent aux besoins d'accompagnement des enfants en situation de handicap les besoins de l'institution scolaire et, surtout, les moyens qu'elle y consentira, notamment en raison de la généralisation des pôles inclusifs d'accompagnement localisés.

avec des temps de travail calculés sur la base minimale de 41 semaines, est visiblement interprétée de façon très diverse d'une académie à l'autre, certaines allant jusqu'à continuer à faire signer des contrats d'un an.

paritaire, confirmant l'accélération de la mise en place d'une école à deux vitesses. « Nous assistons à une stratégie d'une partie de nos élites pour finalement mieux contrôler leur reproduction sociale et lever les derniers obstacles que l'" ancien monde " leur opposait

les finalités et le fonctionnement de l'éducation nationale : enseignement professionnel, baccalauréat, lycée, programmes, tout y passe, sans oublier la sélection imposée à l'accès à l'enseignement supérieur ! Mais qu'on ne s'y trompe pas si les dispositions du présent projet de loi ont été adoptées dans les deux hémicycles, le pays ne les a pas acceptées. La mobilisation dans nos territoires a été inédite et l'opposition conjointe des acteurs de l'éducation comme des parents d'élèves et des élus locaux témoigne d'un mécontentement qui ne s'évanouira pas une fois la loi promulguée. Pour

Marie-Pierre Monier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après plusieurs mois de débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous nous apprêtons à nous prononcer sur la proposition de loi pour une école de la confiance. La CMP a abouti à un accord entre nos deux chambres. Si je me réjouis, avec l'ensemble des membres du groupe socialiste, que le travail réalisé par le Sénat ait permis plusieurs modifications importantes auxquelles nous tenions, ce texte comporte encore des points problématiques sur lesquels je souhaite revenir. Mais, avant toute chose, je veux souligner un point positif majeur, démontrant à mon sens, encore une fois, combien le travail que nous effectuons ici au Sénat, en portant la voix de nos territoires, est d'une grande importance. Je pense bien sûr à la suppression de l'article 6 et fondamentaux, les EPLESF. Ces établissements XXL risquaient d'entraîner des bouleversements profonds dans la structure du système scolaire et auraient eu de lourdes conséquences pour les élèves, leurs familles, les personnels et les territoires, notamment ruraux. Cette suppression est une victoire pour les élus et pour tous les acteurs de la communauté éducative qui s'étaient fortement mobilisés contre Pendant l'examen du texte au Sénat, notre appel à la responsabilité pour sauvegarder nos écoles et, avec elles, nos territoires, avait été entendu par mes collègues. Je me réjouis que nous ayons ensuite su porter cela conjointement, avec la détermination nécessaire. La CMP a fait preuve de sagesse en maintenant cette suppression, et je veux saluer le travail collectif, mené en bonne intelligence et de toute part sur cette question. C'est ce qui permet d'aboutir à ce résultat.

je regrette que les modifications de l'article 4, qui avaient ouvert à toutes les communes la compensation financière liée à l'abaissement de l'âge de la scolarisation obligatoire à 3 ans, aient été supprimées par la CMP :

Malgré quelques apports positifs du Sénat, l'examen du texte par la chambre haute a été marqué par une forte droitisation. Je pense, par exemple, à la suppression des allocations familiales pour les parents d'élèves absentéistes, que nous avions supprimée en 2013 et que le Sénat a réintroduite. Cette mesure aurait pénalisé particulièrement les familles les plus précaires, notamment les familles monoparentales. Fort heureusement, la CMP ne l'a pas conservée.

Pourtant, convaincus que nous aurions pu introduire dans ce texte une autre vision de l'éducation, et animés par la volonté de travailler collectivement sur un sujet aussi important que l'avenir des enfants de notre pays,

Ainsi, malgré la suppression de l'article 6 et quelques autres modifications, le texte sorti du Sénat présentait encore beaucoup trop de similitudes avec le projet de loi d'origine. Il n'est donc pas surprenant que nous retrouvions dans ce texte final, issu de la CMP, un grand nombre de points qui reflètent une vision de l'éducation obéissant d'abord à une logique comptable, qui n'est pas la nôtre. Ce texte ne répond en aucune façon aux véritables problèmes actuels du système éducatif manque de moyens financiers et matériels, la crise des vocations, l'épuisement du personnel de l'éducation nationale et la reproduction des inégalités sociales. Monsieur le ministre, malgré nos mises en garde répétées, vous n'avez pas voulu entendre que l'inscription du devoir d'exemplarité des enseignants, au travers de l'article 1, n'est ni utile ni souhaitable. Cette mention laisse planer, laisse planer, sur l'ensemble des membres de la communauté éducative, une suspicion qui n'est pas de nature à restaurer un climat de confiance. Nous craignons aussi pour l'avenir de l'accompagnement des élèves en situation de handicap : les AESH sont désormais inscrits dans des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les Ce dispositif entérine une mutualisation des moyens qui sera menée au détriment de l'accompagnement personnalisé des élèves et dans des conditions d'exercice très difficiles pour les personnels concernés.

et je le répète : nous ne pouvons accepter de voir se substituer à de nécessaires créations de postes la naissance, l'article 14, d'un nouveau statut incertain et précaire pour des étudiants sans diplôme ni formation pédagogique. se verront confier des missions d'enseignement sans réelles garanties de ne pas se retrouver seuls trop tôt devant une classe. En outre, nous nous inquiétons du rôle qui sera assumé par les missions locales, du fait de l'obligation de formation

Nous ne comprenons pas non plus votre obstination à supprimer le Cnesco. Cette instance fonctionne, avec une grande indépendance d'esprit, notamment grâce à sa composition. Elle met en avant les travaux de la recherche scientifique et permet ainsi de sortir de débats souvent stériles. Les quelques modifications apportées dans la composition de votre nouveau conseil ne changent pas grand-chose sur le fond. Elles illustrent surtout votre politique de reprise en main de l'institution scolaire par le ministère et par vous-même. Malgré les quelques améliorations permises par la CMP, les membres du groupe socialiste et républicain ne peuvent donc pas se satisfaire du résultat obtenu. D'ailleurs, cette CMP est-elle vraiment conclusive ?

deux d'entre elles ont été adoptées : l'une porte sur l'annualisation du temps de service des enseignants, l'autre permet d'associer le chef d'établissement à l'affectation des enseignants. dispositions pour le moins problématiques, et cette manière de les réintroduire doit nous interroger, surtout quand leur auteur est le rapporteur d'un texte sur lequel un compromis a été trouvé Pour en revenir au texte qui nous intéresse aujourd'hui, je réaffirme que le mécontentement des enseignants doit être entendu. S'ils, si elles se mobilisent, c'est bien parce qu'ils et elles tremblent pour l'avenir de notre éducation nationale de loi vient conclure un cycle de réformes, avec la mise en place de Parcoursup, la réforme du lycée, y compris celle du lycée professionnel, et du bac, en passant par les suppressions de postes aux concours et la modification de certains programmes. C'est la défiance qui règne au sein de la communauté éducative : la confiance ne se décrète pas, elle se construit, et ce n'est malheureusement pas le chemin que vous empruntez. Le présent texte s'inscrit donc dans la suite logique d'une réforme de l'enseignement

Je l'ai déclaré à plusieurs reprises : ce choix ne correspond pas à notre vision de l'école de la République. Nous voulons une école qui forme les citoyennes et les citoyens de demain, en leur donnant les moyens de penser par eux-mêmes, une école qui permette de s'extraire du déterminisme social et qui donne le temps à chacune et à chacun de se former suffisamment suffisamment pour pouvoir choisir la vie qu'elle ou il souhaite mener, une école qui est au coeur de la vie des territoires, comme elle le fut sous la III République, grâce à ses « hussards noirs », une école qui soit un véritable lieu d'émancipation et qui permette de croire que, demain, nos enfants auront les outils pour bâtir une société

mais aussi de ses apports majeurs sur la formation des enseignants. Je salue également le dialogue constructif qui a eu lieu avec M. le ministre pendant les débats au Sénat. « Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace », déclarait Jean Jaurès dans son discours d'Albi. C'est proclamer que des milliers d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action ; qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre. défendait une idée de la société et un courage d'esprit que l'école se doit de transmettre ; un idéal, certes, mais qu'il faut toujours et encore cherche à atteindre, en période de crise du lien social. On a pu dire que l'obligation scolaire à 3 ans ne changera pas les choses. Je suis persuadée du contraire : elle fera entrer dans le creuset de l'intégration les enfants de notre pays et fabriquera de la transitionnalité entre la famille et la vie sociale au sein d'un groupe qui, déjà, fait société.

L'obligation de formation jusqu'à 18 ans me paraît être le bon objectif, à la condition évidente de développer les formations d'avenir vers les savoir-faire à la française, la transition numérique, la transition écologique, et de structurer davantage le service public de la formation. Monsieur le ministre, votre objectif est le bon, mais il reste beaucoup de travail à accomplir. Le contrôle de cette obligation ne saurait reposer sur les seules missions locales. L'ensemble des acteurs de la formation tout au long de la vie Nous attendons aussi beaucoup, d'ici à 2022, de la structuration des campus d'excellence dans nos régions, capables de dynamiser la filière professionnelle et de susciter les vocations dans notre pays. Si la formulation du devoir d'engagement et d'exemplarité des enseignants m'a laissé un temps perplexe, je reprendrai les mots prononcés par Ferdinand Buisson, dans son discours du 19 janvier 1910 à la Chambre des députés Laissons à l'instituteur la responsabilité de sa conduite, c'est la meilleure garantie que nous puissions avoir qu'elle soit irréprochable. Le compromis trouvé au Sénat et conservé en CMP a finalement permis de construire en miroir une obligation de respect due aux professeurs, attendue de tous. À la suite d'un amendement déposé au Sénat, l'opinion publique s'est saisie d'une autre question : l'application du principe de neutralité religieuse aux accompagnateurs scolaires, qui a suscité un riche débat. par le Conseil d'État élude à mon sens la question, en posant le principe de non-soumission à la neutralité religieuse auquel le directeur d'école peut déroger par des recommandations au cas par cas. Le bon sens exige de ne plus laisser au directeur la responsabilité de s'exposer et le risque de provoquer des troubles au vu de recommandations qui pourraient être reçues comme une atteinte personnelle. C'est au législateur de prendre cette responsabilité. La règle du cas par cas est, selon moi, trop lâche. Il est urgent d'édicter une règle générale, connue et respectée de tous Si la commission mixte paritaire a écarté cette disposition, elle a retenu l'interdiction des propos prosélytes. Longtemps, la seule disposition de droit interne relative au prosélytisme figurait à l'article 31 de la loi de 1905. L'encadrement juridique du prosélytisme, à géométrie variable depuis plusieurs années, impliquera désormais de porter une appréciation quant aux notions de pression sur les croyances et de tentative d'endoctrinement.

En matière d'évaluation, nous avons regretté la suppression du Cnesco et la disparition de sa fonction de recherche au sein du futur conseil d'évaluation de l'école.

Je pense notamment à l'inscription de l'obligation de formation continue des enseignants, que le groupe du RDSE avait proposée et qui constitue un progrès considérable.

Je pense à la formation dite « continuée », qui est aussi une belle victoire de la chambre haute. Préconisée dans le rapport du Sénat, elle me semble essentielle pour garantir la bonne adaptation des nouveaux enseignants à leur métier. Je pense enfin au dispositif de préprofessionnalisation, qui permet de confirmer le choix du métier d'enseignant avant de présenter le concours. Il s'inspire, lui aussi, des recommandations du Sénat. vous nous avez déjà détaillé un certain nombre de garanties qui entoureraient le dispositif, et qui sont venues me rassurer : un temps de travail limité à huit heures par semaine en établissement, l'accompagnement réel de l'assistant d'éducation par un tuteur, ainsi que la progressivité des missions. Les textes d'application devront en prendre la mesure. Je voterai en faveur du projet de loi pour une école de la confiance, au regard de ses apports pour l'attractivité du métier d'enseignant et parce que je crois à l'extension de la scolarité obligatoire et de l'obligation de formation comme

nous arrivons aujourd'hui au terme de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, après un long travail préparatoire et plusieurs semaines de discussions, parfois passionnées, dans cet hémicycle, comme à l'Assemblée nationale, ainsi que sur le terrain, au contact des acteurs locaux : élus, personnel de l'éducation et, évidemment, parents. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont réussi à s'accorder sur une rédaction commune du texte en commission mixte paritaire,

Je souhaite également remercier, de nouveau, le rapporteur, Max Brisson, et la présidente de la commission, Catherine Morin-Desailly, ainsi que l'ensemble des sénateurs de leur implication dans la conduite de nos débats. En 1870, disait-on, la France avait été vaincue par l'instituteur prussien. L'institution scolaire était effectivement restée un parent pauvre de l'action publique depuis le peu d'enfants allaient à l'école, malgré la loi Guizot de 1833, qui prévoyait l'ouverture d'une école primaire de garçons dans chaque commune. La République s'est donc mise à l'école allemande : l'instruction est devenue obligatoire et le système français s'est doté d'un corps d'enseignants compétents formés dans les écoles normales. Jules Ferry n'invente pas l'école, mais il crée celle de la République et la dote de fonctionnaires aux qualifications et à l'autorité reconnues. « lire, écrire, compter » devient-il une réalité. Un mythe national est né : celui d'un enseignement creuset de la République, porteur de ses valeurs de patriotisme, de laïcité et d'égalité des chances.

Il rappelle le constat de l'enquête PISA : l'école française est peu performante pour les enfants des milieux modestes ; elle accroît les inégalités sociales entre les générations ; elle se contente de comptabiliser les décrocheurs, qui ne sont que trop rarement récupérés pour être remis dans le système. Notons enfin que ce chiffre n'inclut pas les bacheliers qui échouent au début de leur premier cycle universitaire. Nos travaux relatifs au présent texte s'inscrivent dans cette réalité contemporaine. Il était important de le rappeler. Vous-même, monsieur le ministre, avez présenté ce projet de loi comme « une nouvelle étape de cette épopée glorieuse de l'école depuis la fin du XIX siècle ». L'examen de ce texte a été l'occasion pour notre assemblée de jouer pleinement son rôle de représentant des collectivités territoriales, en introduisant un certain pragmatisme, indispensable à la nécessaire application de la réforme sur le terrain. Je pense notamment aux mesures concernant la formation initiale et continue des enseignants, à la composition du futur conseil d'évaluation de l'école, qui sera à même de garantir son indépendance et donc sa crédibilité, ou encore à la lutte contre le prosélytisme et, plus généralement, à la défense des valeurs fondamentales de l'école, qui se trouvent renforcées. Si nous regardons plus en détail le texte final, nous nous satisfaisons également des dispositions relatives à l'obligation d'instruction à 3 ans, même si nous regrettons que l'ensemble des communes ne bénéficient pas d'une compensation financière intégrale, compte tenu Si l'objectif du Gouvernement est louable, le Sénat a très justement prévu, au titre de cette mesure, des aménagements utiles pour les familles et les professionnels. Il en est ainsi de l'obligation d'assiduité en petite section, mais aussi de l'extension à cinq à cinq ans, au lieu de deux, de la dérogation accordée aux jardins d'enfants pour accueillir des enfants d'âge scolaire. Ainsi, l'on pourra faciliter l'adaptation de ces structures au nouveau cadre législatif. Enfin, la CMP a avalisé la position adoptée par le Sénat sur l'article 6. En instituant les fameux établissements publics des savoirs fondamentaux, destinés à réunir école et collège, cet article avait suscité les débats que l'on connaît. Nous nous réjouissons de l'engagement du Gouvernement à approfondir la réflexion sur ce sujet. Le groupe que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui n'est pas en reste concernant les avancées présentes dans le texte. Ainsi, c'est sur l'initiative d'Hervé Maurey et de Catherine Morin-Desailly que les objectifs de l'éducation au développement durable et de l'enseignement numérique prévus dans le code de l'éducation ont été redéfinis et renforcés dans leur ambition, pour faire des enfants des acteurs de la transition écologique et numérique. De même, notre collègue Françoise Gatel a permis que l'État dispose d'un droit de regard sur l'évolution des établissements hors contrat, une fois accomplies les formalités d'ouverture. pense à la suppression de l'article 16, demandée par Jocelyne Guidez afin de rassurer nos infirmiers scolaires. J'ai également en tête plusieurs avancées importantes, que nous souhaitions depuis longtemps, pour l'organisation du temps de travail des enseignants ou encore l'intégration des enjeux territoriaux dans la répartition des moyens.

coupables non pas de réussir, mais de ne pas agir pour autoriser le succès des autres. Trop souvent, l'école ne favorise pas assez de destins communs ; à l'inverse, elle trace des devenirs parallèles. C'est un scandale moral et une faillite économique, contre lesquels nous devons lutter. C'est aussi un péril politique comment une démocratie saine peut-elle durer sur ces bases, en excluant de la réussite toute une partie de la population ? Les statistiques sont malheureusement assez

À l'inverse, les enfants de l'élite réussiront : s'ils n'intègrent pas les meilleurs établissements, ils partiront étudier à l'étranger et auront de bonnes chances de s'en sortir, forts du capital parental. Pour relever les défis du nouveau siècle, la France a besoin de repenser la formation de sa jeunesse. On peut parier qu'elle ne la rendra efficace que si elle la décloisonne, c'est-à-dire si elle s'ouvre à plus de mixité sociale tout en oeuvrant à plus de synergie entre les différents acteurs, agissant de de concert et, oserais-je dire, en confiance. Nous en sommes convaincus : cette lutte pour la mixité sociale et la réussite éducative passent par une plus forte collaboration avec les collectivités territoriales,

vous pourrez compter sur notre sagesse, vous le savez, pour que l'école de la confiance, que nous appelons de nos voeux, continue de faire l'objet d'un véritable travail approfondi, dans un climat apaisé.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, je tiens tout nous voici arrivés au terme d'un processus législatif, avec les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 13 juin dernier. Avant tout, j'adresse mes félicitations à notre collègue Max Brisson, rapporteur, pour la qualité de son travail, ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires qui ont oeuvré de façon collégiale à l'amélioration des dispositions qui s'appliqueront bientôt à l'ensemble de la communauté éducative et des élèves scolarisés en France. sa version finale, ce projet de loi est un texte de compromis, aboutissement de longues discussions au sein des deux assemblées et hors les murs. Il s'articule autour de mesures phares, que les élus de notre groupe ont soutenues. L'abaissement de l'âge obligatoire de scolarité à 3 ans s'inscrit dans un ensemble plus large de mesures visant à réduire les inégalités sociales de réussite scolaire. Le résultat des études PISA, conduites par l'OCDE, traduit la situation alarmante de la France, qui, malgré notre modèle de réussite fondé sur le mérite, compte parmi les pays les plus reproducteurs d'inégalités sociales à la naissance. outre, l'obligation de formation de 16 à 18 ans permettra de mieux lutter contre le décrochage scolaire et d'améliorer l'insertion des jeunes dans la société.

Enfin, l'ouverture à l'international de notre système scolaire se matérialise par le développement prochain des établissements publics locaux d'enseignement international, contribuant à la fois au rayonnement de la France et à la modernisation de notre système scolaire.

qui est extrêmement importante. Je pense notamment à l'introduction d'une formation complémentaire des jeunes enseignants, afin de mieux les accompagner à l'exercice de leurs nouvelles responsabilités ; à l'enrichissement du contenu de leur formation, qui comprendra désormais un volet d'éducation au développement durable encore à l'obligation d'une formation continue pour les professeurs. Le cadre législatif garantissant la laïcité et protégeant la liberté de conscience des élèves au sein des écoles publiques françaises a également été renforcé, ce que nous ne pouvons que saluer. à la possibilité d'aménager l'obligation d'assiduité pour les enfants scolarisés en petite section de maternelle, elle contribuera à l'application en toute intelligence de cette réforme. Nous saluons également l'adoption définitive de certaines propositions introduites par l'Assemblée nationale, notamment la disposition visant à lutter contre le harcèlement scolaire, dont l'actualité nous en rappelle l'urgence

enfin, l'instauration d'une visite médicale à 3 ou 4 ans, pour déceler certains troubles et prévenir les difficultés d'apprentissage. Toutefois, nous regrettons que ces avancées aient eu pour corollaire la suppression de la compensation complète pour les communes participant au financement des classes maternelles privées sous contrat, ainsi que la disparition programmée d'ici à cinq ans des jardins d'enfants, qui avaient pourtant fait leurs preuves. Mes chers

l'année scolaire 2019-2020 s'ouvrira avec l'obligation, et même avec le droit absolu, pour tous les enfants âgés de 3 ans, de suivre une instruction. Par-delà l'aspect symbolique et les questions soulevées par l'application de cette mesure, nous avons tous reconnu l'avancée éminemment sociale que ce changement, voté à l'unanimité par notre assemblée, constituera pour plus de 25 000 nouveaux élèves. En effet, si les 1 000 premiers jours sont primordiaux pour la santé de l'enfant, les premières années sont essentielles dans la capacité d'apprentissage. Elles sont également déterminantes dans la construction des inégalités et du décrochage scolaire. Pour ces raisons, et parce que, de Mayotte jusqu'à la Guyane, en passant par Paris et la Haute-Savoie, la situation sociale, économique et culturelle de nos enfants n'est pas uniforme, il nous fallait consolider le cadre de l'école républicaine et faire de la maternelle une école à part entière. Nos débats ont été riches et ont parfois révélé des désaccords profonds. Nous avons néanmoins parcouru du chemin dans le bon sens et les discussions en commission mixte paritaire se sont rapidement orientées vers un accord. Certaines dispositions auxquelles nous étions radicalement opposés, comme la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme, ont été écartées ; d'autres, au contraire, ont été conservées à la faveur de compromis pertinents, c'est notamment le cas de l'accompagnement financier des communes, de la dérogation temporaire au profit des jardins d'enfants ou encore de la composition du conseil d'évaluation de l'école. Il nous faut donc saluer la volonté du Gouvernement, la sagesse du Parlement, tout particulièrement celle du Sénat, et l'excellent travail accompli par notre rapporteur, Max Brisson. C'est ainsi que l'on arrive à un tel résultat, dont il ne faut pas négliger la portée. Cet accord préserve en effet l'esprit de la politique du Gouvernement en faveur de l'élévation du niveau général des élèves et d'une plus grande justice sociale, tout en préservant les apports du Sénat l'affirmation du rôle du professeur, la dérogation en faveur des jardins d'enfants, la suppression des établissements publics des savoirs fondamentaux, mais également les dispositions spécifiques à l'enseignement en langue régionale ou aux enjeux propres à la Guyane et à Mayotte, ainsi que vous l'avez signalé, monsieur le ministre. de ce texte, qui a suscité de vives inquiétudes- parfois en raison d'imprécisions réelles, le plus souvent à cause de contre-vérités -les clarifications apportées au cours de notre discussion démontrent, s'il en était besoin, l'importance de la navette parlementaire et du Sénat. Personne ne me contredira sur ce point, nos échanges ont été denses, et parfois passionnés ; ils nous ont permis de soulever des questions qui trouveront, j'en forme le voeu, des réponses dans un avenir proche, au travers d'un dialogue nourri avec l'éducation nationale. de la situation des jardins d'enfants. La CMP a réussi à trouver un point d'équilibre en autorisant une dérogation de cinq ans, afin de permettre à ces structures d'entamer une transition favorable. C'est une bonne chose, il ne reste maintenant qu'à engager la discussion avec tous les acteurs et à accompagner les personnels.

Il s'agit d'une décision sage, qui doit renforcer notre volonté d'aboutir à la formalisation d'un véritable statut, lequel sera le fruit, là encore, du dialogue social que le ministère s'est engagé à mener avec les syndicats. S'agissant de l'école inclusive et des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, nous devons garantir à tous les enfants, dans leur diversité, un même accès à l'éducation, en déployant des solutions adaptées.

À cet égard, je me réjouis que ce texte prévoie, d'une part, d'y analyser les effets de l'application de l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire, et, d'autre part, d'autoriser les élus à construire plus rapidement des établissements scolaires du premier degré. Je pense, enfin,

sujet éminemment important pour nos territoires. Une chose est sûre, l'examen de ce texte a pu susciter chez chacun de nous une forme de frustration, tant il nous a menés vers d'autres questions. Vous en conviendrez, mes chers collègues, c'est précisément ce qui fait de l'école un sujet aussi passionnant qu'exigeant.

Monsieur le président, monsieur le ministre,

Il ne s'agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. » Ce projet de loi, monsieur le ministre, peut participer

Il nous faut cependant, comme dans l'esprit de la loi Guizot, qui imposait à chaque commune d'avoir une école publique- nous pourrions ajouter « ou une école privée » -, faire sortir du sommeil cette école du socle commun en menant un débat apaisé avec les maires, les enseignants, les parents et tous les élus.

monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour une école de la confiance a suscité un certain espoir, en raison des difficultés rencontrées par notre système éducatif. Il a aussi provoqué de profondes inquiétudes, chez les élus locaux, les enseignants et les parents d'enfants handicapés, en raison de la création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL. Cette mesure, qui ne figurait pas dans le texte initial, a été introduite en séance publique à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement. Pour ma part, j'insisterai sur les avancées en matière d'inclusion scolaire, lesquelles sont nombreuses, grâce au Sénat, qui a su prendre en compte à la fois les besoins des élèves handicapés et les attentes professionnelles fortes de leurs accompagnants. Je remercie très sincèrement notre rapporteur Max Brisson et la présidente de la commission Catherine Morin-Desailly de leur soutien

Dans ce contexte, le nombre d'enfants handicapés scolarisés a connu une augmentation considérable, de 210 000 en 2004 à 391 000 à la rentrée 2017, entièrement réalisée en milieu ordinaire, comme l'a souligné notre rapporteur.

À cela s'ajoute la multiplication des prescriptions individuelles pour des quotités horaires déterminées qui rigidifient considérablement le système et rendent le métier d'accompagnant peu attractif. Autant d'enjeux auxquels le Gouvernement n'a répondu que très partiellement, en se contentant, d'une part, de créer les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui sont censés être un outil de gestion des ressources humaines et, à ce titre, sont fortement décriés par les d'autre part, de prévoir que les AESH soient recrutés par contrat d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Lors de l'examen du projet de loi par la commission de la culture, plusieurs amendements visant précisément à répondre aux attentes exprimées par les familles et les AESH ont été adoptés. Notre collègue Olivier Paccaud a ainsi présenté un amendement tendant à préciser que les PIAL ne pouvaient pas avoir pour seul objet d'être des outils de gestion des AESH, mais devaient constituer des pôles de ressources à destination de l'ensemble de la communauté éducative, en associant au dispositif les professionnels de santé. Il a également défendu le recrutement conjoint des AESH par l'État et par les collectivités territoriales, afin de favoriser leur emploi à temps complet, ainsi que la prise en charge des élèves en situation de handicap hors du temps scolaire. Notre collègue Philippe Mouiller a, quant à lui, proposé que le retour à une aide individuelle soit possible à chaque instant de la scolarité. Cette disposition utile a malheureusement été supprimée par la CMP. Lors de la séance publique, le texte a été de nouveau enrichi par les apports de plusieurs amendements de notre collègue Philippe Mouiller. Le premier visait à renforcer la coopération entre les professionnels de l'éducation nationale et ceux du secteur médico-social dans l'objectif d'une école plus inclusive, en assurant la présence et l'intervention des équipes médico-sociales au sein des établissements scolaires. tendait à élargir à l'ensemble des établissements et des services médico-sociaux accompagnant les jeunes en situation de handicap la possibilité de s'organiser en dispositif intégré, comme c'est le cas pour les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP. L'appui médico-social au parcours scolaire des jeunes élèves handicapés s'en trouvera facilité. Enfin, s'il n'était pas envisageable de créer un nouveau corps au sein de l'éducation nationale pour y intégrer tous les accompagnants des élèves en situation de handicap, j'ai souhaité, pour ma part, mettre l'accent sur leur formation professionnelle continue. Alors que la demande de suivi individuel ou mutualisé des élèves handicapés explose et que le milieu scolaire ordinaire accueille une plus grande diversité de handicaps, le besoin de formations adaptées s'avère particulièrement aigu, de l'avis même des accompagnants, qui jugent indispensable un renforcement de leur professionnalisation. C'est pourquoi j'ai proposé au Sénat que leur formation professionnelle continue soit fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des élèves. Mes chers collègues, la CMP a maintenu la très grande majorité des dispositions concernant l'école inclusive que nous avions adoptées en première lecture. nous en réjouissons : ce sont de nouvelles avancées pour les enfants, leurs familles et leurs accompagnants, mais aussi pour la société tout entière, avec le renforcement de l'égalité réelle des droits des élèves handicapés. Permettez-moi toutefois d'exprimer un regret : celui d'avoir dû retirer, en CMP, face à des incompréhensions et à des attaques injustifiées, une disposition qui précisait que la scolarisation en milieu ordinaire était un droit, dans la mesure où elle favorisait les apprentissages et permettait de conforter l'enfant handicapé dans ses acquis pédagogiques. Avec cet amendement, il n'était évidemment pas question, pour moi, de mettre en cause le droit à une scolarisation dans un environnement classique, mais plutôt d'éviter que le Gouvernement ne soit tenté de maintenir le statu quo concernant les instituts médico-éducatifs, ou IME, qui souffrent d'un manque cruel de places.

Notre devoir collectif est clair : tout enfant, quelle que soit sa situation personnelle, doit être accueilli dans le système éducatif de la Nation. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, je tiens tout comme chaque fois que nous en avons l'occasion- ce n'est pas rare en ce moment -, nous pouvons nous féliciter que cette commission mixte paritaire ait été conclusive, preuve, si besoin en était, de la vitalité du bicamérisme en France. Puisqu'il s'agit d'un texte qui aura un impact immédiat sur l'organisation scolaire, cela permet, de surcroît, d'envisager une rentrée relativement sereine en septembre prochain, alors que le contexte est aujourd'hui quelque peu tendu. peu tendu. Je veux saluer le travail effectué par notre rapporteur Max Brisson, qui s'est fortement investi sur ce texte, ne ménageant pas sa peine pour faire preuve de pédagogie presque partout en France et même jusqu'auprès de certains ses collègues, collègues, dans un contexte de vives contestations dans le débat public et de mobilisation tant des équipes éducatives que des parents d'élèves et des élus locaux.

l'article 6 , a été supprimée par le Sénat et n'a pas été réintroduite en commission mixte paritaire. Sur ce point, il faut saluer le travail de notre excellent collègue Jacques Grosperrin, qui avait proposé en séance un amendement d'appel, lieu à un débat nourri dans l'hémicycle et,, à un engagement ministériel notable, véritable caution d'un chemin possible vers un consensus en La notion d'exemplarité des professeurs- à laquelle j'aurais, à titre personnel, préféré celle de « neutralité » -a longuement alimenté les débats et vivement inquiété la communauté éducative. Le Sénat n'a pas supprimé cette disposition, mais a souhaité inscrire explicitement à l'article 1 qu'elle allait de pair avec le respect dû par les élèves aux professeurs et avec l'affirmation, dans le droit, de l'autorité de ces derniers. Je me réjouis, par ailleurs, du maintien de l'aménagement temporaire de l'assiduité de l'enfant

sur proposition de la famille et dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, atteint un certain équilibre. Concernant les jardins d'enfants, sénateurs et députés sont parvenus à une rédaction de compromis, qui pérennise ces structures pour un délai de cinq ans. Au-delà des amalgames trop souvent diffusés sur différents bancs, nous souhaitons que cette période leur permette de se reconvertir- ce qui ne sera pas simple -moyennant un accompagnement du ministère de l'éducation. « CMP » peut également signifier « conclusions moyennement positives » ! Ainsi, au sujet des règles de compensation par l'État des charges liées à l'instruction dès 3 ans, je déplore que la majorité gouvernementale soit revenue sur plusieurs dispositions introduites par le Sénat. Le Gouvernement refuse ainsi de prendre en compte la situation des communes qui participaient déjà à la prise en charge partielle des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées, en accueillant des élèves dès 3 ans. Si j'entends l'argument juridique, je regrette que ce biais n'ait pas été suffisamment anticipé. La CMP a retenu la possibilité, pour une commune, de réévaluer les ressources, mais en la limitant aux années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Ce délai est, de mon point de vue, totalement incompatible avec les fluctuations démographiques que peuvent connaître certains territoires. Enfin, je déplore la suppression systématique de toutes les avancées en faveur de la promotion du sport, portées, notamment, par les différents amendements déposés par Michel Savin. D'autres mesures, sans doute davantage dans l'air du temps, comme la sensibilisation au développement durable, ont été privilégiées. Je n'y vois qu'un très mauvais signal envoyé à l'ensemble des acteurs du monde sportif, après les dispositions relatives à l'Agence nationale du sport examinées mardi en séance. Je suis pourtant convaincu, comme bien d'autres, que bien des valeurs sont transmissibles dès le plus jeune âge

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement. Je donne lecture du texte élaboré par la commission

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 15 mai dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun. Cet accord, qui est le fruit d'échanges constructifs avec mon homologue rapporteur le député Dominique Da Silva, devrait nous conduire à voter définitivement cette proposition de loi initiée par le président du groupe La République En Marche de l'Assemblée nationale. Ce texte ouvre la possibilité aux assurés de résilier leur contrat de complémentaire santé à tout moment, passée la première année de souscription, et non plus seulement à chaque échéance annuelle. C'est donc, non pas une complète nouveauté, encore moins une révolution, mais une souplesse supplémentaire, offerte aux ménages comme aux entreprises. L'ambition est à la fois de faciliter la vie des assurés, dans le sillon de plusieurs évolutions législatives récentes dans le domaine des assurances portées par les lois Chatel, Hamon ou Bourquin, mais aussi de renforcer la concurrence sur un marché qui représente, je vous le rappelle, près de 36 milliards d'euros, afin de favoriser une plus grande efficience de ses acteurs. Parce que l'on touche au domaine bien particulier de la santé, cette proposition de loi a suscité des réactions vives et a donné lieu à un large débat au sein de notre commission des affaires sociales, avec des interrogations, notamment, quant à son impact sur les mécanismes de solidarité des mutuelles. Je n'y reviendrai pas en détail aujourd'hui. Il me semble cependant, sans chercher à idéaliser les effets potentiels de ce texte, apporte une contribution utile pour créer les conditions d'un marché plus fluide et pour inciter les opérateurs à proposer de meilleures garanties, aux meilleurs tarifs, pour les assurés. des marges de progression existent. Il nous appartiendra toutefois d'attacher la plus grande attention au suivi de ses effets sur le comportement des assurés, des mutuelles ou des assureurs, ainsi que sur les tarifs des contrats. Au Sénat, les quatre articles formant le coeur de cette proposition de loi, initialement supprimés par la commission des affaires sociales, ont été rétablis en séance publique sur l'initiative de notre collègue Philippe Dallier, pour les articles 1 à 3, et par l'adoption d'amendements identiques déposés en mon nom propre et par le Gouvernement en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur du dispositif.

Cet accord a naturellement été maintenu par la commission mixte paritaire, sous réserve de quelques ajustements concernant les modalités de résiliation des contrats : l'Assemblée nationale avait proposé de largement simplifier ces modalités, mais nous avons rétabli le formalisme de la lettre recommandée dans certaines situations, dans une logique de protection des assurés. mixte paritaire ont principalement porté sur les articles contenant des dispositions que l'on peut qualifier de périphériques par rapport à l'objet initial de la proposition de loi. La CMP a tout d'abord confirmé la rédaction du Sénat pour l'article 3 , introduit par l'Assemblée nationale, qui complète l'information des assurés sur le taux de redistribution des contrats, c'est-à-dire le ratio prestations sur cotisations. Elle a maintenu, en outre, la suppression par le Sénat d'un article inséré par l'Assemblée nationale demandant un rapport sur l'application par les organismes complémentaires des engagements en matière de lisibilité des contrats. Si l'enjeu de transparence est crucial, la portée de l'article restait celle d'une simple demande de rapport. Nous resterons néanmoins très vigilants sur les avancées dans ce dossier, lequel est à l'ordre du jour du comité de suivi de la réforme du reste à charge zéro et fait l'objet d'attentes fortes de la part des assurés. La volonté partagée de recentrer le texte sur son objectif principal a également conduit la commission mixte paritaire à supprimer une disposition, introduite par le Sénat, concernant l'interdiction des pratiques de remboursement différencié par les organismes complémentaires dans le cadre de réseaux de soins. Ce sujet, qui correspond à une position déjà prise par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, trouvera un meilleur véhicule législatif. Les travaux de la CMP nous ont enfin conduits à réintroduire, dans une rédaction moins ambiguë, un article initialement supprimé au Sénat, sur le suivi du déploiement par les organismes complémentaires de services numériques permettant aux assurés, comme aux professionnels et aux établissements de santé, d'avoir un accès en temps réel à leurs droits et garanties. Nous avons partagé l'objectif de sécuriser le tiers payant dans le contexte de l'entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle des contrats. Il n'en reste pas moins que, au-delà des avancées qui pourront être impulsées par les organismes complémentaires, des travaux restent nécessaires, notamment à l'hôpital, pour déployer des logiciels métiers et des interfaces compatibles. Mes chers collègues, le texte issu des travaux de la CMP constitue un excellent compromis. Tout à fait ! Il remplit l'objectif initial de la proposition de loi : mettre en oeuvre la faculté de résiliation sans frais

Merci, est à Mme la ministre. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de m'exprimer devant vous au sujet des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé.

La possibilité de résilier un contrat de complémentaire santé sans frais et à tout moment, au terme de la première année de souscription, est une mesure attendue par les assurés ; elle facilitera leurs démarches et leur permettra d'agir pour leur pouvoir d'achat.

Ce texte s'inscrit dans la continuité des mesures adoptées à la fin de l'année dernière pour répondre à l'urgence économique et sociale et soutenir le pouvoir d'achat des Français. Ainsi, en décembre dernier, les organismes complémentaires ont répondu à la demande du Président de la République en présentant plusieurs propositions pour agir sur les dépenses contraintes des Français, celles auxquelles les ménages ne peuvent échapper. ils ont neutralisé la hausse des tarifs prévue cette année pour les contrats d'entrée de gamme et se sont engagés dans un travail commun pour faire évoluer à la baisse les frais de gestion, qui, je le rappelle, représentent environ 20 % des cotisations collectées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a entendu les remarques formulées par certains parlementaires lors des débats, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Nous n'en suivrons que plus attentivement la mise en oeuvre de la future loi, pour nous assurer qu'elle n'aura pas d'effets négatifs sur l'accès des Français à une complémentaire santé. cette mesure ne devra pas augmenter le coût des primes. Au contraire, l'augmentation de la concurrence qu'elle permet devra inciter les complémentaires à diminuer leurs primes, notamment en réduisant leurs frais de fonctionnement, afin d'attirer ou de garder des assurés. C'est d'ailleurs cet effet qui a été observé dans le domaine de l'assurance emprunteur. Ensuite, la mesure ne devra pas déstabiliser le marché. Conçue pour favoriser la mobilité des assurés désireux de changer de complémentaire santé, elle ne devrait pas bouleverser la situation actuelle, actuelle, la résiliation d'un contrat étant déjà possible à chaque échéance annuelle. Une attention particulière sera portée aux conséquences de cette mesure pour les personnes âgées. Les garanties en termes de mutualisation demeureront inchangées, y compris en faveur des plus vulnérables- j'y serai particulièrement attentive. Les mutuelles et les autres organismes proposant des contrats responsables, qui constituent la quasi-totalité des contrats, ne pourront recueillir d'informations médicales auprès de leurs membres, ni fixer des cotisations en fonction de l'état de santé des assurés. J'y insiste : cette

effet, les personnes âgées sont les plus soumises aux augmentations brusques de cotisations des contrats individuels, et il peut être aujourd'hui difficile pour une personne âgée, souvent non familiarisée avec les nouvelles technologies, de trouver un nouveau contrat dans le délai imparti Les mesures de la proposition de loi bénéficieront aux particuliers, pour les contrats individuels, comme aux entreprises, pour les contrats collectifs. Elles entreront en vigueur au plus tard en décembre 2020 ce délai est évidemment essentiel, puisqu'il permettra la concertation avec les acteurs et surtout la préparation de la mise en oeuvre du texte avec les organismes complémentaires et les professionnels de santé, pour que la mesure se traduise par une vraie simplification pour les assurés. Nous veillerons aussi à ce que les professionnels pratiquant le tiers payant aient accès aux droits des assurés en temps réel, dès lors que les garanties ne couvriront plus nécessairement l'année civile. Enfin, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, le Gouvernement souhaite poursuivre dans un climat de confiance les travaux communs conduits avec les organismes complémentaires depuis le début du quinquennat. Cette collaboration riche a déjà donné lieu à des avancées majeures, comme la réforme du « 100 % santé » : marquant un progrès d'importance dans l'accès aux soins, elle a été construite en liaison étroite avec l'ensemble des acteurs, en particulier les fédérations d'organismes complémentaires.

sur la proposition de loi visant à permettre aux assurés, particuliers comme entreprises, de résilier sans frais et à tout moment, après la première année de souscription, leur contrat de complémentaire santé.

En filigrane, il y a l'idée selon laquelle le renforcement de la concurrence sur le marché des complémentaires ferait baisser le coût des contrats au profit du pouvoir d'achat des ménages.

pour lequel la seule question qui vaille serait celle du calcul des coûts et des avantages pour soi-même, et rien que pour soi-même ! Cette proposition de loi heurte, nous le pensons, le pilier même de notre système de protection sociale : la valeur de solidarité. Elle profitera peut-être à des assurés solvables, jeunes, actifs et bien portants, dans une logique purement assurantielle- des adhérents qui seront encore plus fortement encouragés à individualiser leurs risques en se tournant vers les propositions les moins onéreuses.

L'individualisation du droit triomphe, primant toute logique collective et universelle et venant emboutir le modèle prudentiel français. Des comportements opportunistes, consuméristes ou nomades ne seront pas écartés, même si ce n'est pas là l'essentiel, alors qu'une partie importante des frais de santé pris en charge par les complémentaires correspondent à des dépenses programmables. les gains de pouvoir d'achat des adhérents sont, à notre sens, assez illusoires. L'augmentation du nombre des entrées et des sorties accroîtra le volume et la complexité de la gestion administrative. Il en résultera

... Surtout, aucune réponse n'est apportée aux questions du moment. L'accès aux soins de nos concitoyens s'en trouvera-t-il amélioré ? Non. Les inégalités liées à l'âge seront-elles amenuisées ? Bien au contraire. Les coûts de gestion vont-ils baisser ? Certainement pas. Les actions de prévention menées par nombre de mutuelles seront-elles renforcées ? C'est le contraire qui est à craindre. Le nombre de personnes sans complémentaire

3 A, de charger l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, l'Unocam, de s'assurer du déploiement effectif par les organismes complémentaires des services numériques permettant aux professionnels de santé de vérifier facilement

L'association Inter-AMC, créée en 2015, regroupe tous les acteurs de la sphère complémentaire, y compris les délégataires de gestion, courtiers et opérateurs de tiers payant. Elle propose, depuis la fin de 2016, des services en ligne pour les professionnels de santé de ville. Comme l'IGAS l'a souligné dans un rapport de février 2018, la difficulté tient à l'équipement des professionnels de santé en logiciels compatibles. Il nous aurait semblé plus logique de solliciter cette inspection, qui a déjà réalisé un travail important sur ce sujet, pour suivre l'avancée de la mise en ligne des services pendant une période déterminée.

un virage fort et décisif vers le système beveridgien- universalité, financement par l'impôt, budget indifférencié de celui de l'État

c'est avec une certaine satisfaction que le groupe du RDSE considère ce texte issu d'une commission mixte paritaire conclusive, symbole de vitalité démocratique et d'un travail en bonne intelligence entre les deux assemblées. Alors que la partie semblait, à première vue, mal engagée, compte tenu du texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat- qui ne reflétait pas la position majoritaire de notre assemblée -, les rapporteurs et présidents de commission des deux chambres ont fini par trouver un terrain d'entente, assez proche de la proposition de loi initiale. En ce qui concerne la disposition centrale du texte, la possibilité de résilier une complémentaire santé à n'importe quel moment après la première année de souscription, le groupe du RDSE se réjouit qu'un consensus ait été trouvé en cette mesure, qui entrera en vigueur en décembre 2020, offrira une souplesse supplémentaire aux usagers et, nous l'espérons, une concurrence accrue entre les organismes au profit des Français. Comme il a été rappelé plusieurs fois, les tarifs des complémentaires santé ont augmenté de façon exponentielle à partir de 2010, du fait notamment des frais de gestion, qui représentent aujourd'hui jusqu'à 21 % du coût de la cotisation. Nous ne pouvons nous satisfaire d'une telle situation, dans un domaine aussi sensible que celui de la santé et dans un contexte de vieillissement de la population et d'explosion des maladies chroniques. Pour y répondre, outre la simplification des conditions de résiliation, cette proposition de loi offrira une plus grande transparence aux usagers : les organismes seront contraints de communiquer leur taux de redistribution et le montant de leurs frais de gestion. Les souscripteurs feront ainsi leur choix en connaissance de cause. Nous avons tous reçu des sollicitations nombreuses de mutuelles qui craignent une déstabilisation du secteur en cas d'adoption de cette

Les organismes peuvent, je crois, se rassurer, d'autant que l'utilisation plus fréquente d'une mutuelle par rapport à une assurance habitation rendra sans doute le changement d'organisme plus délicat.

la disparition de l'article, introduit au Sénat, prévoyant l'interdiction des taux de remboursement différenciés pour les réseaux de soins. Ces remboursements différenciés remettent en cause un principe fondamental : à cotisations égales, prestations égales. Néanmoins, nous avons bien compris que cette mesure n'avait pas de lien direct avec le texte initial et constituait, dès lors, un cavalier. Reste que le rapport de force entre mutuelles et assurés doit être rééquilibré, comme l'a signalé notre collègue Stéphane Artano en première lecture. Cette proposition de loi y concourt, dans un contexte de tensions grandissantes entre les pouvoirs publics et les organismes complémentaires. À l'occasion d'une réunion entre tous les acteurs de la réforme du reste à charge zéro, la ministre de la santé elle-même a souligné que les hausses de cotisations avaient rendu la situation difficile pour un grand nombre de Français, et que les augmentations annoncées par le secteur pour l'application du « 100 % santé » n'étaient pas acceptables. Elle a également appelé les assureurs à plus de lisibilité et de modération sur les frais de gestion, point sur lequel cette proposition de loi apporte une première réponse.

Pour les contrats hors assurance vie proposés tant par les sociétés d'assurance que par les mutuelles ou les institutions de prévoyance, y compris les contrats de complémentaire santé, une faculté de résiliation annuelle est déjà prévue, à chaque anniversaire du contrat. Le taux de résiliation annuelle atteindrait 15 % à 20 % en santé et oscillerait autour de 15 % pour les assurances dommages habitation et automobile.

des contrats de complémentaire santé, une fois le premier anniversaire passé. En somme, ces articles opèrent une simplification et une modernisation des modalités de notification d'une résiliation de contrat d'assurance par l'assuré.

par les organismes de complémentaire pour les réseaux de soins, j'y suis favorable, mais je crois que cette mesure doit être approfondie de nouveau ou réétudiée ultérieurement.

Je rappelle que les mutuelles et organismes à but non lucratif sont les premiers acteurs du secteur, avec 51 % de parts de marché. Les sociétés d'assurance représentent 31 % du marché et les institutions de prévoyance, 18 %. L'assurance 18 %. L'assurance complémentaire santé représente 85 % du chiffre d'affaires des mutuelles et 50 % de celui des institutions de prévoyance. En revanche, elle compte pour 5 % seulement de l'activité des sociétés d'assurance.

ce n'est pas contradictoire, mais j'irai même plus loin : les mutuelles et OCAM doivent faire plus d'efforts d'adaptation comme de gestion et être plus proches de leurs sociétaires ; dire cela, selon moi, c'est les servir et les aider à pérenniser ce mode d'organisation. madame la ministre, je réitère mon voeu de voir soumis au Parlement un projet de loi sur la prise en charge de la santé. Si l'accès aux soins et à une médecine de qualité est d'abord assuré par l'assurance maladie obligatoire, qui prend en charge 76,6 % des frais médicaux des Français, les organismes complémentaires d'assurance maladie et assurances privées, facultatives pour la plupart des assurés sociaux,

95 % des assurés, soit la quasi-totalité de la population. Toutefois, la mise en place des contrats collectifs santé et l'essor des surcomplémentaires ont conduit à une prise en charge à trois étages. Ce mode d'organisation complexe me semble contradictoire avec l'objectif politique d'une solidarité exigeante.

part, je crois qu'il serait opportun de définir clairement le niveau de prise en charge relevant uniquement de la solidarité nationale et de laisser à chacun la liberté d'adapter précisément sa couverture en fonction de ses besoins

Nous savons que la hausse des cotisations, de 30 % en dix ans, est source d'insécurité financière pour les foyers les plus démunis. Aussi le groupe Les Indépendants - République et territoires se félicite-t-il du succès de la commission mixte paritaire, qui a abouti, le 15 mai dernier, à un texte de compromis. Il est vrai que nous aurions pu aller plus loin : d'une part, en accélérant l'entrée en vigueur de cette réforme, prévue en décembre 2020 d'autre part, en maintenant l'interdiction de la pratique des remboursements différenciés par les mutuelles, mesure que j'avais proposée à la commission des affaires sociales, qui l'avait adoptée. Le désaccord entre les deux assemblées à ce sujet n'est pas nouveau, puisque la dernière remise en question des réseaux de soins par le Sénat date du projet de Nous persistons à penser que cette pratique va à l'encontre de la liberté de choisir son praticien de santé et augmente les inégalités individuelles de remboursement des soins. Nous le savons, le secteur le plus touché est l'optique, où un tiers des complémentaires fonctionnent avec des réseaux fermés, imposant à leurs adhérents d'aller chez les praticiens partenaires et de choisir certaines marques, certains modèles de verres ou de lentilles correctrices. Il est regrettable que la commission mixte paritaire ait rejeté la proposition du Sénat de supprimer cette pratique. Cette mesure concrète et attendue était complémentaire de celles contenues dans la présente proposition de loi. Notre groupe et, je l'espère, l'ensemble du Sénat resteront engagés pour faire aboutir cette évolution législative souhaitable. L'objectif principal de la proposition de loi est néanmoins préservé. Notre groupe est très favorable à la résiliation infra-annuelle des complémentaires santé, associée au renforcement de la lisibilité des contrats. Cette clarification permettra à chacun de comparer plus facilement la qualité de la protection offerte par chaque société et, ainsi, de souscrire avec une plus grande liberté de conscience le contrat

la proposition de loi sur sa disposition initiale : la possibilité de résilier après un an d'adhésion, à tout moment et sans frais, les contrats de complémentaire santé. Même si je regrette la suppression de la mesure introduite par le Sénat pour mettre un terme à la pratique des remboursements différenciés par les réseaux de soins, je la comprends

de loi prévoit également de compléter l'information des assurés sur les taux de redistribution des contrats, c'est-à-dire le rapport entre les prestations versées et les cotisations encaissées. Il vise un objectif de transparence sur les contrats de complémentaire santé auquel le groupe Les Républicains ne peut que souscrire. Je tiens à vous rappeler, quitte à me répéter- mais la pédagogie est affaire de répétition -, que les frais de gestion de la sécurité sociale s'élèvent à 4,5 %, alors que ceux des complémentaires santé sont, en moyenne, de 20 % à 25 % et peuvent atteindre 42 %.

est de constater qu'il découle de ces différentes réformes un marché de la complémentaire santé très administré, dont le cadre réglementaire et fiscal est pour le moins sophistiqué. Pour autant, ce marché reste peu protecteur pour nos concitoyens qui n'entrent dans aucun dispositif spécifique : les jeunes, les inactifs, les retraités. Nous avons déjà vu des secteurs entiers, que la puissance publique n'a pas su réguler, connaître une transformation radicale sous l'effet d'une concurrence accrue. Cela ne sera sans doute pas le cas pour les complémentaires santé du seul effet de ce texte, mais donner de la souplesse revient, à nos yeux, à renforcer la marge de manoeuvre des assurés. L'évaluation de l'impact de cette mesure est difficile à évaluer : baisse des coûts et hausse du pouvoir d'achat pour les uns, risque de nomadisme et de démutualisation pour les autres. Les débats ont été nourris, à la fois au sein de la commission des affaires sociales et dans l'hémicycle. Il me semble peu probable que cette disposition bouleverse l'économie des contrats collectifs des grandes entreprises. Celles-ci ont évidemment les moyens de sélectionner au mieux l'organisme qui leur convient et de gérer leur calendrier de résiliation, par ailleurs enserré dans un processus de négociation collective. Pour les plus petites entreprises comme pour les adhésions individuelles, le texte apporte une souplesse supplémentaire par rapport à la possibilité de résiliation annuelle. il reste encore des efforts à faire en termes de lisibilité des contrats. Ce n'est pas tout de donner aux Français la possibilité de changer de complémentaire santé ou de mutuelle ; encore faut-il leur donner les moyens de décrypter Ce texte ne répond donc pas à lui seul aux enjeux du secteur des organismes de complémentaire santé, qui restent considérables. À titre personnel, je souhaite considérables. À titre personnel, je souhaite que la sécurité sociale se réapproprie l'ensemble des besoins de santé de base essentiels à nos concitoyens, conformément aux objectifs de ses fondateurs. Mais aujourd'hui, nous sommes bien loin d'une telle réforme systémique qui, je l'espère, viendra malgré tout rapidement. Dans l'immédiat, la grande majorité du groupe Les Républicains votera en faveur de la possibilité offerte aux assurés, après douze mois d'affiliation, de résilier un contrat de complémentaire santé à tout moment. à vous remercier Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après quelques atermoiements, la droite sénatoriale a largement soutenu le principe de la résiliation sans frais des contrats des complémentaires santé à n'importe

sur laquelle les députés de votre parti s'étaient abstenus. Cette convergence pour vanter les mérites d'une plus forte concurrence sur le fameux marché des complémentaires santé ne nous a pas convaincus du bien-fondé de la résiliation des contrats en cours

Depuis la crise de 2008 et l'application de la directive européenne dite Solvabilité 2, les mutuelles sont obligées de disposer d'un montant minimal en euros pour garantir la solvabilité de l'établissement en cas de krach. Cette obligation ne peut pas être correctement respectée si, dans le même temps, les adhérents peuvent résilier à tout moment leur contrat, y compris après un an d'adhésion. Cette volatilité des adhérents est contraire au droit européen, mais également au principe de solidarité des membres d'une mutuelle. Nous faire croire qu'accroître la concurrence sur le marché des complémentaires santé diminuera les tarifs des contrats, en s'appuyant sur l'exemple de l'assurance automobile, nous semble pour le moins inadapté. Les principes mutualistes prévoient l'absence de sélection des adhérents, l'égalité de traitement, la transparence et la solidarité entre mutualistes. Le principe d'annualité des cotisations est en outre un élément du modèle économique permettant de ne sélectionner ni le risque couvert ni la personne. Ces principes trouvent leur traduction dans la comptabilité interne des mutuelles avec, d'un côté, des cotisations stables, et, de l'autre, des prestations qui sont supérieures pour les moins bien-portants et, au contraire, inférieures pour les bien-portants. Ce mécanisme solidaire dans lequel les plus jeunes cotisent le plus souvent pour les plus âgés fonctionne malgré une taxation à 14 % des contrats et l'obligation de solvabilité à hauteur des fonds propres.

Comment prétendre, dès lors, comme le fait le Gouvernement, qu'il s'agit de redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français ? Actuellement, la concurrence entre les organismes complémentaires est déjà très forte en période de fin d'année civile. Il est à craindre que la résiliation en cours d'année entraîne une concurrence exacerbée en permanence et une augmentation des frais de gestion pour financer les frais de publicité. Toutes vos réformes amplifient la marchandisation de la santé,

des sociétés d'assurance à but lucratif et renforcer les mastodontes de la « bancassurance », afin de faire primer le fonctionnement assurantiel sur la logique de solidarité. Ce projet va à l'encontre des objectifs qu'affiche votre gouvernement, madame la ministre, puisqu'il amplifiera le renoncement aux soins d'un public toujours plus large, d'où l'opposition résolue de notre groupe, qui continuera à dénoncer le désengagement de l'État du financement de la sécurité sociale. En effet, c'est bien là le fond du problème. La solution pour empêcher tous ces renoncements aux soins, toutes les inégalités que votre gouvernement amplifie, c'est le 100 % sécurité sociale ! Et ne nous dites pas que ce n'est pas possible : les financements pour y parvenir existent, notre groupe en a fait maintes fois

avant tout, je tiens à remercier mon collègue et ami, Michel Amiel, rapporteur de ce texte, pour la qualité du travail réalisé dans des conditions bien particulières. Cette proposition de loi s'inscrit dans le mouvement engagé par la réforme du « reste à charge zéro » sur les soins dentaires, optiques et auditifs. Elle s'inscrit dans une action globale menée par le Gouvernement pour diminuer les coûts et lutter contre le renoncement aux soins. Pour que cette action soit globale, nous devions nous emparer d'un nouveau volet : le coût de la complémentaire santé. Nous devions l'adapter aux besoins de nos concitoyens. C'est pourquoi la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, donne la possibilité aux assurés de résilier sans frais leurs contrats, et ce à tout moment à l'issue de la première année de souscription. En donnant davantage de liberté aux adhérents, elle rend ce marché plus concurrentiel. C'est le moyen le plus efficace pour atteindre des objectifs concrets et immédiats simplification des démarches, une amélioration du pouvoir d'achat des ménages la réduction des dépenses contraintes pesant sur les adhérents. Et tout cela sans remettre en cause ni la solidarité entre les assurés ni la pérennité des mutuelles qui, nous le savons, ont souvent des coûts de gestions élevés, lesquels coûts sont souvent évoqués, mais qu'il est indispensable de rappeler. Ainsi, selon l'UFC-Que Choisir, les montants des cotisations santé ont augmenté de 47 % au cours de la dernière décennie. Il s'agit d'une hausse significative quand on sait que l'inflation n'a progressé, quant à elle, que de 14,2 % sur la même période. Quant aux frais de gestion, ils ont crû de 30 % depuis 2010, deux fois plus vite que les remboursements. Cette année, pour la première fois, les coûts de gestion des complémentaires santé dépasseront ceux de l'assurance maladie, qui représente pourtant 78 % des soins fournis Avec l'adoption de ce texte, l'économie pour les consommateurs pourrait atteindre 1 milliard d'euros par an. La majorité du Sénat s'était déjà intéressée à ce sujet et proposait de taxer lesdites mutuelles à cette hauteur. Tout à fait ! À la ponction systématique des entreprises, nous préférons un libéralisme bien régulé.

Il a fallu une semaine de réflexion et le dépôt d'amendements de rétablissement, proposés par notre collègue Philippe Dallier, pourtant membre de la commission des finances, pour que la loi retrouve son essence. Ces amendements, rappelons-le, étaient quasiment identiques aux deux amendements proposés, l'un par le rapporteur, l'autre par le Gouvernement. Ayant retrouvé son architecture, la proposition de loi pouvait poursuivre son cheminement et être adoptée par la grande majorité des membres Les deux textes des assemblées étant désormais quasi similaires, la commission mixte paritaire a concentré ses travaux sur les dispositions périphériques qui permettent d'améliorer cette loi. J'en citerai quelques exemples. Le texte entérine la simplification et la modernisation des modalités de notification d'une résiliation. Il rétablit l'obligation de résiliation par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un certain nombre de situations exposées spécifiquement à des risques de contentieux.

Par ailleurs, le texte prévoit de confier à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'Unocam, la mission de s'assurer du déploiement des services numériques par les organismes complémentaires avant l'entrée en vigueur du présent texte. Il s'agit là de la réintroduction de l'article 3 A dans une rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. En ce qui concerne les informations communiquées par les organismes complémentaires dans le cadre des contrats responsables et la date d'entrée en vigueur du droit à résiliation, du droit à résiliation, le texte prévoit de conserver la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Vous l'aurez compris, cet accord constitue un excellent compromis. Le texte est le fruit d'échanges constructifs et devrait nous conduire à voter définitivement cette proposition de loi. Sans grande surprise, le groupe La République En Marche votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. La discussion Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Merci,